Bien entendu, pour que cette liberté s'exerce dans le respect de chacun, elle doit être encadrée par la loi. À cet égard, la pandémie que nous traversons oblige à définir de nouvelles règles. Il s'agit de mesures barrières. À ce titre, il est peu compréhensible que les policiers ne bénéficient pas d'équipements de protection pour les contrôles. D'ailleurs, l'éloignement des individus les uns des autres en limitant la liberté d'aller et venir ne peut être que transitoire. Les Français ont bien compris cette nécessité et ont très majoritairement fait preuve de civisme. Il faut garder à l'esprit que l'objectif de ces règles est de garantir la liberté et la sécurité de chacun. Avec le déconfinement, des interrogations demeurent pour plusieurs situations au-delà de 100 kilomètres : des étudiants finissent leur année et vont souhaiter rentrer chez leurs parents des personnes âgées sont isolées depuis trop longtemps et ont besoin d'être soutenues par leurs proches. Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs, mais rappellent que la vie familiale des Français n'est pas une option. Il ne faudrait pas sacrifier la liberté de tous par crainte de l'irresponsabilité de quelques-uns.

de la liberté de circulation. À partir du 11 mai, les Français pourront sortir librement dans la rue, sans attestation. Néanmoins, nous voulons évidemment éviter que le virus ne se propage

un but sanitaire. Nous ne doutons d'ailleurs pas que nos concitoyens respecteront une fois de plus cette règle, comme ils ont respecté les règles qui s'appliquaient pendant le confinement. Cette règle de l'interdiction des déplacements au-delà de 100 kilomètres du domicile connaîtra effectivement des exceptions. Vous avez rappelé les motifs prévus, à savoir des motifs familiaux ou professionnels impérieux, qui seront définis. Le Premier ministre s'exprimera demain sur les conditions de mise en oeuvre de cette mesure et nous donnerons un certain nombre de cas dans lesquels les déplacements seront permis. Néanmoins, je me réfère à ce qu'ont dit le Premier ministre et le Président de la République : nous ferons surtout appel au civisme de nos concitoyens. Nous comptons beaucoup sur la

Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où les parents d'élèves s'inquiètent, où les directeurs d'école redoutent cette date du 11 mai et ses nombreuses inconnues, où les maires s'interrogent sur leur capacité à répondre à la lourdeur écrasante des protocoles qui leur sont imposés, il est temps que le Gouvernement rassure en envoyant des signes clairs et forts. Trop d'interrogations demeurent sur la question des moyens. Je pense aux masques, au gel ou encore aux concours financiers pour soutenir les communes et les intercommunalités qui mettraient en oeuvre les activités périscolaires que vous avez dénommées « sport, santé, civisme et culture ». À ce propos, nous souhaiterions une réponse précise : quel protocole s'appliquera pour ces activités périscolaires ? un protocole spécifique ou un protocole scolaire ?

et aux directeurs d'établissement l'assurance que, en appliquant des consignes qu'ils n'ont en rien décidées, ils ne sauraient être poursuivis en cas de nouvelles contaminations. Il s'agit d'un préalable essentiel si l'on veut garantir un climat de confiance indispensable à cette rentrée scolaire. Ma question est claire : soutiendrez-vous cette disposition afin que la sortie du confinement souhaitée ne devienne pas une date redoutée ? La parole

parce que le virus fait peur, parce que beaucoup d'inconnues subsistent encore à la fois sur l'impact médical, sur la réalité de ce virus et sur ses modes de transmission. Par ailleurs, après une si longue période de confinement, reprendre une vie normale, même prudemment, même progressivement, a forcément quelque chose d'inquiétant.

qui s'interrogent sur les bonnes décisions à prendre. Quelquefois, mais à titre infiniment subsidiaire, ils se posent aussi des questions sur la mise en cause de la responsabilité qui pourrait être la leur.

J'ai indiqué ici même, à la tribune, lundi, à l'occasion de la présentation du plan de déconfinement, que ces questions étaient importantes et qu'il fallait les traiter sérieusement. J'entends parfaitement que le Parlement, dans son pouvoir souverain, puisse essayer d'apporter des améliorations.

trop facilement et trop systématiquement attaquée dans des cas où ils ne peuvent être tenus pour responsables. Je crois que ce dispositif est bon. S'agissant de la réouverture des écoles, c'est l'État qui prend la responsabilité de les rouvrir. C'est l'État qui a fermé les écoles et c'est l'État qui décidera de les rouvrir. Il s'agit bien d'une responsabilité de l'État. Sans doute faut-il préciser, s'agissant de la responsabilité civile ou de la responsabilité pénale,

Sans doute. Mais atténuer, monsieur le sénateur, la responsabilité d'une catégorie de décideurs ou même de tous les décideurs ne me semble pas une bonne idée. Je le dis comme je le pense, en étant conscient que ma réponse peut

la responsabilité des décideurs, nous ne rendrions pas service à notre pays et nous ne redonnerions pas confiance à nos concitoyens. Je me permets donc de dire clairement que je ne m'inscris pas du tout dans une logique d'atténuation de la responsabilité.

réplique, et à lui seul ! Certes, monsieur le Premier ministre, c'est l'État qui prend la responsabilité, mais vous ne pouvez pas méconnaître que ce sont les maires qui seront à la manoeuvre, y compris lorsqu'il s'agira,

de la meilleure façon, il importe plus que jamais de renouer le lien de la confiance. C'est cette confiance qui permettra toutes les formes de réussite ! La parole monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, les gens du voyage entament chaque année, dès la mi-mai, une traversée du pays en direction du littoral atlantique ou du sud méditerranéen. Cela concerne jusqu'à 25 000 personnes. intercommunale), compétents en matière d'accueil, sont extrêmement inquiets en cette période de crise sanitaire. En effet, les « grands rassemblements » sont des pèlerinages de foi auxquels il pourrait être difficile de renoncer. Monsieur le secrétaire d'État, ces mouvements de population conduiraient à d'inévitables catastrophes que les élus de proximité auraient à gérer, en plus du reste ! Nous nous trouvons très souvent, dans cette période de crise, placés en situation d'urgence. C'est pourquoi je souhaite être rassurée sur le fait que les risques liés à ces déplacements ont été anticipés

les gens du voyage respectent, comme tous les Français, les mesures prévues à cet effet, avec l'appui des préfets et des responsables associatifs des gens du voyage, avec lesquels nous sommes d'ailleurs en discussion permanente. Dans le cadre de la période qui s'ouvrira à compter de lundi, deux mesures vont concerner les gens du voyage, comme l'ensemble des Français : celle que j'ai évoquée à l'instant en répondant au sénateur Joël Guerriau, et qui interdit les déplacements au-delà de 100 kilomètres

que nos concitoyens gens du voyage respecteront cette interdiction. Je puis vous dire que mes services sont en contact avec les associations représentatives des gens du voyage et que nous discutons d'ores et déjà de ces sujets. Nous continuerons, bien évidemment, à dialoguer avec eux. le civisme dont ils ont fait preuve, comme tous les Français, pour le respect des mesures de confinement nous laisse augurer qu'il n'y aura pas de non-respect des règles que nous allons fixer à compter du 11 mai. Je puis vous le garantir, madame la sénatrice,

Le Parlement comme le Gouvernement sont au chevet de l'économie française. Nous avons déjà voté deux lois de finances rectificatives, qui reposent sur des outils principaux nous connaissons bien désormais. L'activité partielle, qui concerne six salariés sur dix, le fonds de solidarité pour les petites entreprises, les prêts garantis pour sauvegarder la trésorerie et les prises de participation lorsque les grandes entreprises sont menacées : tels sont les quatre principaux piliers de cette action. Nous savons que l'urgence commande d'agir parce que des secteurs sont très menacés. Je pense, bien sûr, à l'hôtellerie, à la restauration et au tourisme, qui font l'excellence française. Je pense aussi aux grands noms ou aux gens moins connus du secteur culturel, qui sont une âme de notre pays. À cet égard, les annonces du Président de la République aujourd'hui vont dans le bon sens et sont de nature à rassurer un secteur véritablement en péril.

allons procéder à une annulation totale de charges entre le 15 mars et le 15 juin pour l'ensemble des secteurs hôtellerie, restauration, tourisme, art et spectacle, culture, sport, et ce pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés.

Les industriels du secteur estiment que la baisse du trafic aérien mondial va affecter non seulement la solvabilité des compagnies aériennes, mais aussi celle des avionneurs et des motoristes. C'est la chaîne d'approvisionnement, représentant 80 % du coût d'un avion, qui sera le plus durement impactée. Les pertes de compétences pourraient être irréversibles pour les industriels de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Les observateurs s'accordent à dire qu'à moyen ou à long terme le marché repartira et que l'industrie aéronautique rebondira. Il convient donc de prendre en compte le risque d'arrivée d'acteurs étrangers, qui viendraient acheter les savoir-faire et compétences qu'il faut parfois dix ans à acquérir sur certains postes, affaiblissant ainsi durablement les avionneurs et les motoristes français et européens. Le plan de soutien du Gouvernement aux compagnies aériennes est accueilli favorablement par les industriels de la filière. Mais encore faut-il alimenter positivement le secteur en permettant de renforcer les commandes, tant en avions dont la flotte devra être renouvelée avec des modèles plus respectueux de l'environnement, qu'en commandes publiques pour la défense nationale. Seuls ces investissements permettront d'alimenter positivement toute la chaîne de production, qui compte de nombreuses PME et ETI (entreprises aujourd'hui fortement fragilisées. Je sais que M. le ministre de l'économie et des finances réunit cet après-midi le comité stratégique de filière. C'est pourquoi, afin de ne pas perdre ce domaine d'excellence industriel où chacun dépend de l'autre, je complète les termes du courrier adressé par mon collègue Alain Chatillon et cosigné par les quinze parlementaires de la Haute-Garonne. Madame la secrétaire d'État, ne serait-il pas important dans cette phase intermédiaire que la France appuie le lancement de nouveaux programmes ambitieux au niveau européen, soutenus par des avances remboursables ? Très bien

nous nous sommes assurés qu'ils avaient bien enclenché les mesures d'urgence, notamment le chômage partiel, qui est la première réponse pour conserver les compétences extraordinaires dont nous disposons dans l'aviation. Vous avez raison de le souligner, il faut parfois dix ans

à la fois d'accompagner l'approvisionnement en équipements de protection et de s'assurer que les protocoles sanitaires sont mis en place dans les meilleures conditions, non seulement dans les grands groupes, ce qui est évidemment le plus facile à réaliser, mais également sur l'ensemble de la filière, dans les PME et les ETI.

des écoles le 11 mai. Cette annonce a suscité de l'espoir. Il restait quatre semaines pour construire et réussir ce plan de déconfinement. Cependant, à quelques jours de cette date, ce sont plutôt incertitude et colère, parfois bien légitime, qui s'expriment dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, les élus locaux sont tous volontaires pour faire vivre le service public dans leur territoire, service public garant de l'égalité républicaine. Mais ils ne sont pas volontaires pour assumer les responsabilités qui ne sont pas les leurs et pour lesquelles ils ne disposent pas de moyens. Ils refusent ainsi d'être demain les coupables, celles et ceux qui, inévitablement, seront pointés du doigt parce que votre décision de rouvrir les écoles le 11 mai les invite inévitablement à rouvrir les cantines, les transports scolaires et, dans quelques semaines, les internats. Ils seront ainsi pointés du doigt parce qu'ils seront responsables de la propagation du virus dans leur territoire. Monsieur le Premier ministre, un protocole sanitaire a été présenté lundi. Vous l'avez lu, nous l'avons lu. Ce protocole sanitaire est souvent contradictoire, mais, surtout, il est inapplicable dans la plupart des écoles de notre République. En période de crise, l'heure n'est pas à faire comme l'on veut l'heure est à assurer partout l'égalité républicaine. Monsieur le Premier ministre, qu'entendez-vous faire d'ici au 11 mai pour assumer vos responsabilités et donner les moyens aux élus locaux de les appliquer ?

vous évoquez d'une certaine manière le désengagement de l'État, qui renverrait la responsabilité, notamment celle de la réouverture des écoles, sur les maires. Vous dites en même temps que, dès lundi dernier, mon collègue Jean-Michel Blanquer a diffusé un texte qui pose le cadre sanitaire et le cadre d'accueil des élèves à partir des recommandations du conseil scientifique. Ce texte a fait l'objet d'une très large concertation avec l'ensemble des associations d'élus. Ce protocole sanitaire fixe donc un cadre précis : les écoles n'ouvriront pas si elles ne sont pas en mesure d'assurer suffisamment de sécurité. Mais l'État ne se désengage pas : il a été clairement précisé qu'il fait confiance aux acteurs qui sont les plus proches du terrain et qu'il accompagnera les communes. Vous demandez en quelque sorte qu'il soit dès lors possible d'inscrire dans un texte de loi une atténuation de la responsabilité

faut soit une faute délibérée, soit une faute caractérisée. C'est la raison pour laquelle il me semble difficile, sauf à préciser la loi, ce à quoi je me suis montrée ouverte et ce à quoi travaillent actuellement, je crois, vos collègues de l'Assemblée nationale, d'aller très au-delà. D'ailleurs, je me permets de faire remarquer ceci : si nous décidions quelque chose pour les élus locaux, en raison du principe d'égalité devant la loi pénale, c'est aussi pour l'ensemble des décideurs qu'il faudrait le faire, à savoir les élus locaux, les décideurs publics, mais aussi les chefs d'entreprise et les décideurs privés. Madame la garde des sceaux, je ne dis jamais « en même temps » ; vous avez donc certainement interprété mes propos. La question n'est pas là. Vous me parlez de droit pénal, je vous parle de ce qui s'exprime aujourd'hui parmi l'ensemble des élus locaux de notre pays. Vous voulez assimiler l'ensemble des décideurs locaux. Eh bien, oui, assimilons-les jusqu'au bout ! Mais, en tout état de cause, à partir du 11 mai, ce sont eux qui auront la responsabilité d'expliquer aux populations pourquoi les écoles sont ouvertes ou fermées et non vous.

Mais les questions ne sont pas l'apanage de la classe politique : ce sont les Français qui s'en posent, ne sachant plus à qui les adresser. Lundi, monsieur le Premier ministre, vous nous avez présenté le plan de déconfinement, et c'est peu dire que nous sommes restés sur notre faim, avec plus de questions que de réponses : priorité donnée à l'exigence de santé ou à la reprise économique ? sécurité sanitaire des enfants ou libération des parents pour retourner travailler ? masques « priorisés » pour les soignants, mais inutiles pour les citoyens, qui, finalement devront obligatoirement en porter dans les transports de la santé), mais encore bien peu usités pour préparer le déconfinement ? distanciation physique quasi impossible dans les transports aériens, urbains scolaires, mais plages et forêts interdites de fréquentation ? Monsieur le Premier ministre, les questions sont nombreuses. Elles sont d'ailleurs le carburant nécessaire au bon fonctionnement de notre démocratie et du débat parlementaire. Mais, alors, pourquoi certains exigent-ils un impossible unanimisme en qualifiant d'« irresponsables » ceux qui expriment doutes, critiques ou oppositions ? Vous n'êtes pas sans avoir observé à quel point le sens des responsabilités a prévalu, ici, lors de l'adoption des différents textes qui nous ont été soumis : deux lois d'urgence, deux lois de finances rectificatives. Nous Nous vous avons accordé beaucoup de moyens pour agir contre cette pandémie désastreuse, mais la démocratie ne doit pas être une victime supplémentaire du Covid-19 ! J'en viens à ma question : acceptez-vous, monsieur le Premier ministre, de tenir compte du rôle du Parlement, majorité et opposition, et d'agir demain pour définir les conditions détaillées du déconfinement sans forcément avoir recours aux ordonnances qui le contournent, celles-ci ayant déjà été largement utilisées quand l'urgence l'exigeait

Mais, à la vérité, lorsque vous me demandez si le Gouvernement est disponible pour répondre aux questions et disponible pour entendre ce que lui disent les représentants de la Nation, la réponse est évidemment « oui ». Pour tout vous dire, je me permets je me permets de m'étonner que vous puissiez en douter, franchement. Nous avons eu ici des débats sérieux, dignes, qui n'étaient pas d'ailleurs nécessairement consensuels ; mais, après tout, les débats servent à cela, et vous l'avez rappelé. Mais je ne crois pas que quiconque puisse dire que le Gouvernement aurait refusé de répondre à des questions, ne serait pas resté disponible, n'aurait pas respecté les commissions du Sénat, n'aurait Que vous ne soyez pas d'accord avec toutes les réponses, je peux l'entendre, c'est normal, c'est la démocratie ; mais ne laissons pas croire, monsieur le président Éblé, à nos concitoyens qu'il y aurait, d'un côté, ceux qui portent la voix vivante de la démocratie et, de l'autre, un gouvernement qui ne voudrait pas l'entendre, parce que cela ne correspond pas à la vérité.

un équilibre, mais vous savez pertinemment que, si nous donnons la priorité à l'une en oubliant l'autre, nous risquons d'avoir de très mauvaises nouvelles.

Nous devons donc reprendre la production, nous devons donc reprendre la vie sociale, nous devons donc reprendre l'école, parce que, sinon, c'est la catastrophe ! Nous savons aussi que, si nous allons trop vite, par enthousiasme, par imprudence, en privilégiant cette fois-ci la reprise sur la sécurité sanitaire, nous risquons, dans ce cas-là, d'avoir de très mauvaises nouvelles sanitaires. Pourquoi, monsieur le président, présenter les choses comme si nous avions délibérément choisi une priorité par rapport à une autre ? Nous essayons justement- ce qui n'est pas facile -de préserver l'équilibre entre ces deux principes. C'est un chemin de crête, c'est vrai, avec deux à-pics vertigineux.

Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » J'avoue, sans polémique aucune, qu'en cette période de prédéconfinement j'ai parfois des difficultés à comprendre toutes les mesures et stratégies, ce qui, forcément, génère de la crainte. Je souhaiterais évoquer en particulier la vie sur le littoral, ainsi qu'un point précis concernant le secteur agricole. La vie sur le littoral du Pas-de-Calais et sur les littoraux de France est rythmée en ce moment par de graves soucis économiques ; mais je retiendrai trois sujets. Premièrement, le secteur de la pêche, même si des aides conjoncturelles sont partiellement actées, craint de ne pas les voir les voir arriver suffisamment tôt pour encaisser le choc et s'inquiète de son avenir quant à l'aboutissement des mesures de chômage partiel. Deuxièmement, la question migratoire. Je soulève ici l'incompréhension des élus locaux et des habitants de la ville de Calais. Malgré les moyens d'accueil mis en place par l'État, le confinement n'est pas respecté par les migrants. Il y a là un vrai sujet d'incompréhensions et de tensions. Troisièmement, le sujet de la réouverture des plages et des espaces de promenade proches du rivage. L'apparition du classement en couleurs inquiète et crée de la confusion. La confiance sur ce sujet, j'en suis convaincu, viendra de l'action qui sera menée entre les préfets et les maires des sites concernés. Des espaces immenses sur le littoral ne me semblent pas plus vecteurs de la contagion que des forêts ou des parcs et jardins. Vous savez comme moi que nous aurons du mal, aux beaux jours, à maîtriser les affluences, et je prône, au plus vite, la concertation pour la mise en place de dispositifs locaux encadrés, qui permettront une réouverture rapide. Pouvez-vous nous donner des perspectives encourageantes sur ces sujets ? Encore un point d'incompréhension, maintenant, sur la politique agricole. L'Union européenne n'a-t-elle pas mieux à faire aujourd'hui que d'introduire un accord de libre-échange avec le Mexique, dont le calendrier est une pure maladresse ? C'est évident ! Quels que soient les termes de cet accord, la crise sanitaire a fait prendre conscience que notre souveraineté dans les domaines tant sanitaire qu'alimentaire était essentielle, favorisant de fait les circuits courts. Pourquoi envoyer ce message contradictoire en cette période troublée ? Quelle est la position du Gouvernement à ce sujet ? M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous comprendrez que, dans le temps qui m'est imparti, je ne pourrai répondre à l'ensemble des questions sur lesquelles vous interpellez le Gouvernement, dont certaines touchent à la politique agricole ou à la politique économique. Je vais néanmoins répondre à

Pas-de-Calais. Je vous confirme effectivement qu'un certain nombre de migrants ne respectent pas les mesures de confinement, ce qui nous a conduits à lancer- ce dont vous avez été forcément informé -plusieurs opérations que nous appelons « opérations de mise à l'abri

Un déconfinement progressif va cependant commencer lundi prochain, provoquant chez les Français beaucoup d'inquiétudes quant à la situation sanitaire mais aussi économique et sociale qui pourrait les impacter durablement. Le choc économique va être très violent, plus encore dans les secteurs d'activité qui ne pourront pas reprendre le 11 mai, comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel et d'autres encore. À période exceptionnelle, mesures économiques et sociales exceptionnelles. Pour permettre la survie de milliers de TPE-PME, qui ont besoin de visibilité, il est indispensable d'annuler leurs charges. J'ai noté que vous alliez en déterminer les modalités, auxquelles nous serons attentifs. Il s'agit non pas de générosité, comme le Gouvernement a pu le dire, mais de nécessité. Je veux aussi insister sur les salariés actuellement en chômage partiel, plus de 11 millions de personnes. Si la mise en activité partielle permet d'amortir le choc, elle risque d'aller au-delà du 11 mai pour les secteurs qui ne peuvent redémarrer. Le groupe socialiste et républicain souhaite, dans tous ces cas, le maintien du chômage partiel dans sa forme actuelle, sans dégressivité et au-delà du 1 juin. Des effets pervers se profilent pour les droits à la retraite de certains salariés, notamment les moins bien rémunérés d'entre eux, dont l'indemnité de chômage technique n'est pas soumise à cotisations sociales et n'ouvre donc pas de droits. Cela concerne les salariés aux contrats courts ou encore ceux qui font de petits volumes horaires et qui n'atteindront pas les 600 heures de SMIC pour acquérir quatre trimestres de cotisation. Ma question est simple et j'attends une réponse claire allez-vous modifier le dispositif actuel pour que la période de chômage partiel soit prise en compte et puisse donner lieu à des trimestres cotisés pour tous les salariés ? La parole

nous avons pris la décision suivante : je présenterai demain en Conseil des ministres une disposition législative permettant l'acquisition de droits à la retraite de base pendant les périodes d'activité partielle. Cette mesure permettra de mieux protéger les salariés

Elle est durable, évolutive et parfois imprévisible. Qu'en avons-nous déduit ? Que la bataille à conduire doit être collective, mais ordonnée. Qu'avons-nous constaté ? Que les gestions territoriales sont efficaces quand elles réunissent, autour du préfet, l'ensemble des acteurs locaux dans un modèle de qui a pour objectif de résoudre les questions. C'est ce que nous avons vu tout particulièrement dans le Morbihan, en Ille-et-Vilaine et encore ailleurs. Mais nous avons aussi vu des pilotages déficients parce qu'ils étaient éparpillés,

l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté vient d'informer le préfet, par circulaire, de son intention de recruter plus de 120 standardistes pour assurer le suivi et le logement de personnes ayant été en contact avec un cas

des remerciements que vous adressez à l'administration territoriale de l'État, au corps préfectoral, bien sûr, mais aussi à l'ensemble des services de l'État. Je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler que j'en ai moi-même été membre pendant plus de vingt ans de ma vie, ce qui a été un grand honneur. un grand honneur. Christophe Castaner et moi-même sommes très flattés de voir la façon dont nos services gèrent cette crise totalement inédite sur l'ensemble du territoire national. Je parle bien sûr des services des préfectures, des sous-préfectures, et de l'ensemble des services de l'État sur les territoires. Les préfets ont donc des compétences

pleine et entière. Je veux vous rassurer sur un point, s'il le fallait encore. Tous les soirs, le ministre de l'intérieur, en ma présence, réunit l'ensemble des préfets de région et des préfets de zone pour discuter de ces sujets. à nous, une fois par semaine, les directeurs d'ARS justement pour nous permettre de coordonner cette action. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même participe à certaines de ces réunions et donne les impulsions nécessaires. Comme l'a dit le Premier ministre, comme l'a également dit le Président de la République, le moment venu,

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. L'annonce de l'ouverture des écoles le 11 mai prochain suscite encore beaucoup d'incompréhension et d'inquiétude chez les maires. L'État s'appuie très largement sur les élus locaux pour mettre en oeuvre ce dispositif censé être opérationnel dans quelques jours. Ce délai est d'autant plus difficile à tenir qu'un grand nombre de questions concrètes n'ont pas obtenu de réponse. Les maires sont contraints à des choix qui peuvent être lourds de conséquences sur la santé de leur population. C'est aussi le cas des chefs d'entreprise. La question de la responsabilité juridique doit donc être rapidement clarifiée. Pourtant, une fois encore, le Gouvernement a refusé les propositions faites par le Sénat pour répondre à l'inquiétude des maires. Il faut maintenant remédier à cette situation en faisant valider par la préfecture les protocoles établis par les maires. Cette protection juridique est indispensable pour qu'ils puissent agir sans être accusés de fautes qu'ils n'auraient, qu'ils À la question de leur responsabilité s'ajoute celle de la légitimité. En effet, 86 % des communes ont élu au premier tour des municipales un conseil complet. Il est souhaitable que les nouvelles équipes puissent être installées rapidement afin de disposer de la légitimité politique nécessaire. La levée du confinement ayant lieu le 11 mai, peut-on prévoir l'élection des nouveaux maires à une date proche de celle-ci, en respectant bien entendu les règles sanitaires indispensables ? Je vous demande donc, monsieur le Premier ministre, si, d'une part, vous envisagez d'encadrer strictement la responsabilité juridique des maires et si, d'autre part, l'installation des équipes municipales est envisageable à partir du 11 mai.

toutefois, comme vous, qu'il est probablement nécessaire, dans un objectif de réassurance, de clarifier ce cadre juridique dans le contexte très particulier de cette pandémie. Pour autant, je ne pense pas que la solution retenue par le Sénat soit la meilleure. En supprimant la possibilité d'engager la responsabilité pénale de certains décideurs pour une faute caractérisée, le texte qu'il a adopté pourrait donner le sentiment

en droit pénal français. » C'est faux ! Pour notre démocratie, et je suis certaine que vous partagez ce point de vue, il serait délétère de laisser penser que nous souhaitons organiser l'impunité des décideurs dans une période où l'exigence de responsabilité est si essentielle.

Herzog, pour la réplique. Nous savons que ces questions se poseront de nouveau en septembre. Au-delà des écoles, les maires sont sollicités pour l'ensemble du déconfinement et il est donc urgent et nécessaire que ces problèmes juridiques soient réglés rapidement afin de les soutenir au mieux dans leurs fonctions. Nous en

soir : Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire je tiendrai les présidents de groupe politique informés de l'évolution « météorologique », pour que nous puissions adapter nos travaux dans les meilleures conditions. Je n'ignore pas qu'un certain nombre de collègues parcourent de nombreux kilomètres en voiture pour venir jusqu'ici, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Il n'est pas mauvais que nos concitoyens mesurent ce qu'est le travail au quotidien de parlementaires qui entendent que la démocratie vive. Personne ne